monsieur le président,

La séance est reprise. Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement.

Je rappelle que, en raison de l'inaction de l'administration depuis de nombreuses années, ce stock de demandes est substantiel, les plus anciennes remontant à 2009.

Cette rétroactivité aurait pour effet de faire tomber l'ensemble des demandes d'octroi initial de permis de recherches, soit quarante-deux demandes, ainsi que les trois demandes d'octroi initial de concession qui ne relèvent pas du droit de suite. Le Gouvernement nous demande d'adopter une disposition rétroactive, ce qui est contestable sur le plan des droits acquis et de la sécurité juridique, au surplus sans que nous en connaissions véritablement le champ d'application effectif ni les conséquences financières pour l'État.

La prolongation récente du permis « Guyane maritime » serait-elle la seule exception et, si oui, sur quels critères vous êtes-vous fondé pour établir cette unique exception et pour exclure l'octroi d'autres permis ? Je pense en particulier aux deux permis de recherches concernant les deux autres zones situées au large de la Guyane. Sur ce point, nous n'avons pas non plus d'évaluation, même approximative, des indemnisations que l'État devra verser. Or celles-ci sont certaines, puisque la loi reviendra sur les effets légitimement attendus de ces demandes, pour lesquelles le Gouvernement lui-même nous a rappelé que le droit en vigueur ne lui permettait pas de motiver des décisions expresses de rejet : il y a donc bien un droit qu'une loi rétroactive viendrait remettre en cause, ouvrant ainsi un droit à indemnisation. Pourrait-on au moins savoir si ces indemnisations potentielles seront de l'ordre de la dizaine de millions d'euros, de la centaine de millions d'euros, voire davantage ? Je précise que l'État a déjà été condamné à verser plusieurs millions d'euros d'astreintes,

La commission des affaires économiques du Sénat a restreint l'application de l'article 1 prévoyant l'arrêt progressif de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures aux demandes de titre déposées au 6 juillet 2017, en excluant les demandes en cours d'instruction. Afin de préserver l'esprit et l'efficacité du projet de loi, il convient d'appliquer ces dispositions aux demandes en cours d'instruction, eu égard à leur nombre- demandes de titre d'exploration et quatorze demandes de titre d'exploitation au 1 septembre 2017. En effet, une telle dérogation viderait

entre les demandes de titre, sauf celles pour lesquelles une décision de justice est passée en force de chose jugée, enjoignant ainsi à l'administration de délivrer le titre ou d'autoriser sa prolongation. Il avait pour objet de solder le stock de demandes en cours dans les délais les plus brefs possible après l'entrée en vigueur du projet de loi. L'article 2, tel qu'il a été adopté par la commission des affaires économiques du Sénat,

les mots « demandes en cours d'instruction » ne soient interprétés comme se référant aussi à la phase d'instruction des requêtes et appels devant la juridiction administrative et n'ajoutent ainsi implicitement, à l'exception

signifierait, d'une part, revenir sur les effets légitimement attendus des demandes déposées- le Gouvernement lui-même reconnaît que le droit antérieur ne lui permettait pas de les rejeter les rejeter -, et, d'autre part, sanctionner les demandeurs en raison de l'inaction de l'État au cours des dernières années- je rappelle que les demandes les plus anciennes remontent à 2009 -, ce dernier ayant préféré garder le silence plutôt que de prononcer des décisions explicites de rejet qu'il aurait été bien en peine de motiver Là aussi, nous avons recherché un point d'équilibre entre l'exigence de sécurité juridique et l'objectif affiché du Gouvernement d'un arrêt de ces activités à l'horizon 2040. Seules les demandes déposées au plus tard le 6 juillet 2017, soit la date d'adoption par le Gouvernement de son plan Climat comportant l'annonce de « la sortie progressive de la production d'hydrocarbures sur le territoire français à l'horizon 2040 », seront concernées, ce qui évitera tout effet d'aubaine pour les demandeurs. En revanche, l'encadrement du droit de suite, en vertu duquel la durée d'une concession ne pourra dépasser le 1 janvier 2040, sauf si la rentabilité de l'opération exige d'aller au-delà, sera applicable y compris aux demandes en cours d'instruction.

de ce projet de loi. Quant aux demandes qui ont été déposées mais qui ne créaient pas de droit, ce sera éventuellement en contentieux qu'elles seront jugées, selon le droit en vigueur,

Monsieur Labbé,

Mme Primas a parlé avec justesse de la parole de l'État. Or la parole de l'État, c'est la COP21

Nous sommes face au mur et, comme je l'ai déjà dit en commission, si nous ne posons pas maintenant un acte politique fort, dans vingt ans,

Nous proposons cette évolution du droit pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous considérons que ces dispositifs contraignent trop fortement la puissance publique, qui doit conserver la maîtrise de sa politique énergétique et minière.

il nous semble important que le législateur puisse faire évoluer le droit, surtout si celui-ci n'est plus en phase avec l'urgence, reconnue par nos concitoyens, de changer les pratiques en matières énergétique et environnementale. Nous devons faire évoluer le droit

d'intérêt général est ici clair et bien identifié ; il ne fait aucun doute. Il convient dès lors de faire évoluer le droit. Il est possible, dans ces conditions, de remettre en cause des droits acquis, comme l'indique la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Une phase d'indemnisation des concessionnaires sera bien sûr nécessaire, ne nous le cachons pas, mais notre avenir et celui de nos enfants sont à ce prix. lesquelles nous demandons la suppression de ce droit de suite, qui fait primer des intérêts économiques particuliers sur l'intérêt commun et celui de notre planète.

Nous considérons que si seul le titulaire d'un permis exclusif de recherches d'exploration peut obtenir une concession en vue de l'exploitation, l'État ne doit pas, par principe, être tenu d'octroyer une concession sur les gisements exploitables. Nous en reviendrons ainsi à l'esprit de la loi, qui veut que le droit de suite soit un simple droit de non-mise en concurrence, et non un droit automatique

Pour ce faire, nous proposons de soumettre les permis concernés par les dispositions de l'article L. 132-6 du code minier à une enquête publique de toute nouvelle concession lié à la mise en oeuvre du droit de suite. Un tel amendement a déjà été discuté à l'Assemblée nationale. D'autres groupes présentent des amendements similaires. Il a été répondu aux députés qui, en défendant un amendement sur cette question, faisaient également entendre la voix des ONG, que l'enquête publique était déjà prévue par l'article par l'article L. 132-3 du code minier, ainsi que par l'article 26 du décret n° 2006-648, qui prévoit que « toute demande d'exploitation doit faire l'objet d'une enquête publique et être accompagnée d'une notice environnementale Cependant, cette enquête et ces notices environnementales n'ont en réalité aucune portée, les concessions ayant été systématiquement octroyées en raison du caractère automatique, dans les faits, du droit de suite. de l'enquête publique dans le projet de loi vise donc à limiter le caractère automatique du droit de suite et à laisser à l'administration une possibilité effective de refuser certains permis, si cela est nécessaire eu égard aux conclusions de l'enquête publique. Si vous nous dites qu'une telle modification n'est pas nécessaire, car il s'agit déjà du droit positif,

fasse l'objet d'une évaluation environnementale. Il vise ainsi à compléter l'article L. 132-6 du code minier, qui consacre le droit de suite et dont je rappelle les termes : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 142-4, pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci. Le titulaire d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. » Nous proposons, pour encadrer ce droit de suite quasiment automatique, de compléter cet article par un nouvel alinéa ainsi rédigé Préalablement à sa délivrance, la demande d'octroi de concessions est soumise à une évaluation environnementale, en application de la section 2 du chapitre II du titre II du livre I du code de l'environnement. Cette évaluation porte sur les incidences environnementales de l'exploitation du périmètre du périmètre sollicité ainsi que sur les effets notables de la manière dont le demandeur compte procéder. » L'amendement n° 26 rectifié, présenté

à la vérification des exigences définies pour toute autre concession. Nous souhaitons donc que le code minier soit plus précis. Il est nécessaire d'indiquer clairement que la délivrance d'un titre minier d'exploitation dans le cadre du droit de suite doit être assortie de l'obligation de réactualiser les données relatives aux capacités financières et techniques du demandeur.

de droit, et la possibilité de prolonger une concession telle qu'elle est prévue. Cet amendement constitue donc une remise en cause manifeste des droits acquis, qui ouvrirait droit à des indemnisations considérables. Il va bien au-delà de ce que prévoit le texte actuel. La commission émet un avis défavorable, ainsi que sur l'amendement n° 29 rectifié.

rectifié semble lui aussi totalement satisfait par le droit en vigueur, qui dispose, d'une part, que nul ne peut obtenir de permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières adéquates, d'autre part et surtout, qu'il en est de même pour l'attribution d'une concession ou d'une autorisation d'exploitation relativement

et pas simplement les hydrocarbures, je propose d'aborder le sujet en 2018, à l'occasion de la refonte du code minier. L'avis

Il en est de même pour l'enquête publique, qui est déjà prévue. Rappelons aussi que tous les travaux, dont les forages, sont soumis à une étude d'impact et à une enquête publique. Il est vrai que les rares concessions demandées sont souvent accordées, mais ce n'est pas systématiquement le cas.

d'ores et déjà que nul ne peut obtenir un titre minier s'il ne possède pas les capacités techniques et financières nécessaires. De surcroît, mes services, au sein de l'administration centrale et en régions,

de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures, cet article prévoit que la durée de la prolongation d'un permis exclusif de recherches en cours d'instruction soit calculée à compter de l'entrée en vigueur de la décision de prolongation, et non pas à partir de la précédente période de validité du permis.

économiques d'un amendement de la rapporteur, Mme Lamure. Le droit actuel dispose que la prolongation d'un permis exclusif de recherches prend effet à la date d'expiration de la précédente période de validité. Compte tenu de retards constatés dans l'instruction et l'octroi des prolongations de permis, la commission fait observer que certaines prolongations octroyées n'avaient en réalité aucun intérêt. C'est la raison pour laquelle elle propose que, lorsque dans l'attente d'une prolongation de son titre le titulaire d'un permis exclusif de recherches ne poursuit pas ses travaux, la durée de cette prolongation soit calculée à compter de l'entrée en vigueur de la décision de prolongation. L'objectif est clair

Je le rappelle, ces prolongations sont pourtant de droit. Elles ont souvent été accordées bien après l'expiration de la période de validité du permis et peu de temps avant celle de la nouvelle période demandée, ce qui, dans la plupart des cas, leur a fait perdre tout intérêt. Pour répondre à ces situations, le présent article prévoit que la durée de la prolongation soit calculée à compter de l'entrée en vigueur de la décision de prolongation. Cet article nous paraît parfaitement justifié. J'ajoute que, contrairement à ce qui a été indiqué, il appartient bien au législateur

lorsque l'explorateur a fait une demande de prolongation, mais n'a pas mis en oeuvre ce que l'on appelle la « survie provisoire » de son permis, qui lui permet de poursuivre les travaux sans attendre la décision explicite sur la prolongation. cet article excède, selon nous, le champ du présent projet de loi, puisqu'il concerne les permis relatifs à la recherche de toutes les substances de mines, et pas simplement les hydrocarbures. Dans le cas des hydrocarbures, l'application de ses dispositions conduirait à à prolonger notablement la durée de vie des permis, sans cohérence, une fois encore, avec l'objectif d'une cessation d'activité à l'horizon de 2040. Par ailleurs, la possibilité d'accorder la prolongation exceptionnelle jusqu'à trois ans d'un permis de recherches d'hydrocarbures, qui est autorisée par l'article L. 142-2 du code minier, permet déjà à l'État de prendre en compte des situations particulières, instruites au cas par cas, justifiant d'augmenter la durée de validité d'un

Cet article introduit par mes collègues de l'Assemblée nationale a été modifié au Sénat en commission. Sa rédaction mérite aujourd'hui d'être précisée sur plusieurs points.

peuvent être transférées, et pas les installations d'exploitation et d'exploration, tel un puits d'exploitation par exemple. Or l'objectif est bien de pouvoir transférer l'ensemble : il nous paraît important de lever le doute. De plus, en cohérence avec la procédure d'arrêt de travaux, ce transfert doit être approuvé par l'autorité administrative, comme c'est d'ailleurs le cas pour les installations hydrauliques.

pour toutes les installations non nécessaires au nouvel usage lorsqu'ils souhaitent les transférer à l'État, alors qu'ils devraient le faire pour un transfert à toute autre personne publique ou privée, en vertu de l'alinéa 3. La nuance est de taille ! Pour lever cette ambiguïté, nous proposons de supprimer les alinéas 4 et 5, déjà satisfaits par l'alinéa précédent.

ce nouvel article ouvre la possibilité de convertir ou de céder à d'autres personnes publiques ou privées les installations d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures en vue d'autres usages du sous-sol. La commission des affaires économiques du Sénat a complété cet article en prévoyant que l'État puisse décider le transfert à son profit de tout ou partie des droits ou obligations liés à l'activité minière, pour faciliter la conversion des sites miniers après l'arrêt de l'exploitation des hydrocarbures. Nos amendements visent à ce que, dans le premier comme dans le second cas, les collectivités territoriales puissent être associées aux décisions de reconversion des sites miniers.

Enfin, le II supprime la possibilité introduite par la commission d'un transfert à l'État, à son entière discrétion, des droits et obligations associés à l'ancienne activité minière. La commission y est défavorable.

et L. 153-15, peuvent être transférées. Il est également nécessaire de préciser que ce transfert doit être approuvé par l'autorité administrative. Enfin, il n'est pas souhaitable que l'explorateur ou l'exploitant soit exonéré de la procédure d'arrêt de travaux miniers pour toutes les installations non nécessaires au nouvel usage lorsqu'il souhaite notamment les transférer à l'État, alors qu'il devra s'y conformer en cas de transfert à toute autre personne publique ou privée,

Gontard, sur l'article. Le présent article aborde un point très sensible : le traitement des hydrocarbures non conventionnels, c'est-à-dire les gaz et huiles de schiste, les bitumeux, les gaz de couche, les gaz et pétrole de réservoir compact. Il est nécessaire d'être très précis dans la définition de ces hydrocarbures. national de la transition écologique, le CNTE, le 23 juillet dernier. Nous regrettons que le Gouvernement ait suivi l'avis du Conseil d'État et préféré l'approche de la loi de 2011, ne visant que les techniques utilisées pour l'extraction, et faisant abstraction de la nature de l'hydrocarbure. Cette approche nous semble incomplète. L'expérience de la loi de 2011 nous a bien montré que la seule prise en compte des techniques utilisées n'était pas suffisante, d'autant que ce mécanisme se fonde uniquement sur un système d'autodéclaration du détenteur du titre, présumant donc la bonne foi des déclarants. L'expérience récente n'est pas encourageante. Sur seize permis visés, seuls trois ont été abrogés. Les détenteurs ont ainsi mentionné ne pas utiliser la fracturation hydraulique. Cela signifie tout simplement que treize permis sont aujourd'hui dormants et concernent des hydrocarbures non conventionnels, contrairement à ce qui a pu être affirmé dans l'étude d'impact. La différence entre hydrocarbures non conventionnels et conventionnels n'étant pas précisément définie, il est fortement probable que d'autres permis de recherches ou d'exploitation concernent en réalité pour partie des hydrocarbures non conventionnels. Il est indispensable d'agir au regard des graves préjudices écologiques que l'exploration ou l'exploitation de ces hydrocarbures non conventionnels engendrent. Il convient de définir un dispositif efficace pour ne plus permettre l'exploitation de ces hydrocarbures. Nous présenterons donc deux amendements visant à sécuriser ce dispositif. Le premier reprend la définition des techniques interdites proposée par la commission du développement durable de l'Assemblée nationale. Le second vise à soumettre l'ensemble des détenteurs de titres miniers à une nouvelle déclaration, seul moyen d'assurer une prise en compte réelle de l'évolution législative par l'ensemble des détenteurs de titres miniers. Pour autant, nous considérons que ce système présente encore des failles, puisqu'il repose une nouvelle fois sur la seule bonne foi des concessionnaires. Il est donc fort probable que nous ayons besoin à terme d'établir une définition claire des hydrocarbures non conventionnels.

l'examen de cet article 3 pour donner l'éclairage d'un élu d'un territoire directement concerné par la question des hydrocarbures non conventionnels, souvent dénommés gaz de schiste. Pour l'Ardèche, comme pour d'autres départements tels le Gard, la Savoie, la Haute-Savoie ou l'Isère, où a été détectée la présence de schistes bitumineux, il est primordial que la loi interdise de façon explicite la recherche et l'exploitation de tous les hydrocarbures non conventionnels, et ce quel que soit le mode d'extraction. D'abord, celle-ci sera forcément complexe, donc coûteuse, et sa rentabilité ne sera assurée qu'avec le maintien de cours relativement élevés. Or, qui peut prédire aujourd'hui quel sera le cours de ces matières premières dans les décennies à venir ? Ensuite,

en cas de forage profond, en raison des nombreuses failles qui le parcourent et qui jouent un rôle important dans le cheminement des eaux souterraines. Or les ressources de ce territoire, et de ceux qui l'entourent, proviennent principalement d'un tourisme qualitatif fondé sur ses atouts géologiques, en particulier le thermalisme et les activités nautiques dans les gorges de l'Ardèche. des nappes phréatiques, comme celle qui a été constatée en Pennsylvanie en 2013, venait à se produire, les conséquences seraient tout simplement catastrophiques. Ce serait un désastre pour ce tourisme vert qui attire des millions de personnes venues profiter

composé de routes départementales étroites, essentiellement montagneuses, créant un trafic ingérable et dangereux, facteur de nuisances inconciliables avec le modèle économique de nos territoires. Miser sur une énergie déclinante et sur un non-sens économique serait une injure faite à nos enfants. Le gaz et le pétrole ne s'extraient qu'une seule fois, alors que les dommages qu'ils causent sont, eux, irréversibles. L'avenir de nos territoires

Pour autant, peut-on dire qu'il comporte de réelles avancées ? Je pense que nous restons dans le même schéma que celui de la loi de 2011 : ce n'est pas l'exploration-exploitation des hydrocarbures non conventionnels qui est interdite, mais simplement une technique

C'est la situation vécue à Montélimar, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Si de nombreux acteurs environnementaux semblent avoir accepté une définition des hydrocarbures non conventionnels liée à la technique d'exploitation, nous aurions préféré une définition directe de ces hydrocarbures,

il s'agit de la technique de fracturation hydraulique, déjà interdite par la loi Jacob de 2011, ou « de toute autre méthode ayant pour but de conférer à la roche une perméabilité Monsieur le ministre, nous pensons que faire porter l'interdiction sur des techniques plutôt que sur la nature même des hydrocarbures non conventionnels n'est pas de nature à garantir sur le long terme l'interdiction de l'exploration et de l'exploitation de ces hydrocarbures tout à fait spécifiques.

dont l'extraction est source de graves dommages pour l'environnement. C'est pourquoi cet amendement vise à interdire « la recherche et l'exploitation des huiles ou gaz de roche-mère, c'est-à-dire des hydrocarbures liquides ou gazeux qui sont emprisonnés au sein d'une formation de roche non poreuse et dont l'extraction nécessite de fracturer ou de fissurer cette roche par quelque

En effet, le code minier ne différencie pas hydrocarbures conventionnels- pétrole, gaz -et non conventionnels- pétrole et gaz de schiste, de couche ou de roche. Il se borne à interdire la fracturation hydraulique, qui n'est pas la seule technique d'exploitation des hydrocarbures non conventionnels, sans même la définir ... Le projet de loi initial en restait là, mais l'Assemblée nationale, en commission, a proposé une définition précise et complète des techniques utilisées pour l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels. Cette rédaction a été modifiée en séance, sur proposition du Gouvernement, pour viser « toute autre méthode ayant pour but de conférer à la roche une perméabilité ». Cette définition manque de précision et de rigueur scientifique, car toutes les roches présentent

dès la publication de la présente loi, avec l'extraction d'hydrocarbures non conventionnels, dont les ravages écologiques, aux États-Unis ou au Canada par exemple, ne sont plus à démontrer.

qui vise à mieux décrire les techniques qui sont utilisées pour explorer et exploiter les hydrocarbures non conventionnels piégés dans des roches non perméables. Cette définition, qui est peut-être discutable sur le plan scientifique, nous semble préférable à celle figurant à l'amendement n° 48 rectifié, dans la mesure où elle couvre bien toutes les techniques non conventionnelles et ne comporte pas le risque de s'appliquer aux techniques conventionnelles sans danger pour l'environnement. Quant à l'amendement n° 70 rectifié, il repose sur une autre approche consistant à viser des types d'hydrocarbures plutôt que des techniques. Au surplus, l'amendement introduit les notions nouvelles

lorsqu'il s'agit de manipuler des concepts scientifiques qui ne font pas consensus. J'ajoute que nos collègues députés ont ouvert des débats qui n'avaient pas lieu d'être en pratique, puisque l'interdiction de la fracturation hydraulique, combinée aux pouvoirs que la police des mines confère déjà à l'État, nous prémunit déjà contre tous les risques de recours à des techniques non conventionnelles sur le territoire national. La commission émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements. Quel est l'avis du Gouvernement ?

est à Mme le rapporteur. Par souci de clarté, le texte de la commission a codifié dans le code minier les dispositions de la loi Jacob de 2011. Cette codification a été opérée « à droit constant » par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale, afin qu'il ne puisse nous être reproché d'en profiter pour revenir sur tel ou tel point de la loi. Cet objectif de clarification n'ayant pas été contesté, le présent amendement prévoit d'aller au bout de la démarche de simplification en supprimant uniquement des dispositions nouvellement codifiées : les mesures transitoires prévues en 2011, qui n'ont par définition plus lieu d'être.

L'article 3 du projet de loi, qui codifie la loi du 13 juillet 2011, prévoit que le fait de procéder à un forage suivi de fracturation hydraulique de la roche sans l'avoir déclaré à l'autorité administrative dans le rapport précisant les techniques envisagées est passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

de toute autre méthode ayant pour but de conférer à la roche une perméabilité. Au regard des difficultés d'articulation de ces deux sanctions, le présent amendement procède à leur alignement sur la peine prévue à l'article L. 512-1 du code minier, qui sanctionne également d'autres

et non les seuls demandeurs, devront, si nous adoptons cet amendement, justifier auprès de l'autorité administrative qu'ils n'utilisent pas une méthode interdite par le présent article, qui comporte une définition plus large que celle de la loi de 2011. L'adoption garantirait ainsi que les détenteurs actuels de permis ne puissent plus employer aucune méthode de fracturation de la roche ou de stimulation, hydraulique ou autre.

au vu de l'impact environnemental de ces techniques, mais également dans une optique de cohérence de ce projet de loi, il nous semble essentiel de garantir que l'interdiction de ces techniques qui visent à altérer la perméabilité de la roche soit bel et bien respectée par tous.

d'un rapport démontrant l'absence de recours aux techniques interdites. Même si une telle obligation n'aura d'autre effet que d'alourdir inutilement la charge administrative pour les titulaires

Nous proposons, au travers de cet amendement, d'interdire aux sociétés et à leurs filiales ayant leur siège social en France de pratiquer la délocalisation en exploitant les hydrocarbures non conventionnels non conventionnels hors du sol national. Nous souhaitons ainsi renforcer la responsabilité sociale et environnementale des entreprises dans la globalité de leurs activités. Cette responsabilité, si elle ne valait que sur sol national, ne serait que partiellement respectée et peu contraignante pour des sociétés dont l'activité s'exerce principalement à l'étranger.

Nous ne souhaitons pas, en présentant cet amendement, nous poser en « législateur universel », reproche qui avait été adressé à notre ancien collègue Michel Billout en 2011, lorsque notre groupe avait déposé un amendement similaire

? Cet amendement tend à interdire aux sociétés ou à leurs filiales ayant leur siège social en France d'utiliser des techniques dites non conventionnelles dans le cadre de leurs activités hors du territoire national. Une telle interdiction, si elle devait être étendue hors des frontières nationales, ne saurait être fixée par la loi française, mais devrait nécessairement être arrêtée arrêtée au plan européen ou international. En outre, si la France l'adoptait unilatéralement, les sociétés concernées pourraient alors avoir intérêt à déplacer leur siège social hors de France pour contourner la mesure. En conséquence, l'avis est défavorable.

Comme le souligne l'étude d'impact jointe au projet de loi, les activités d'exploration et de production d'hydrocarbures représentent pas moins de 1 500 emplois directs et 4 000 emplois indirects sur le territoire national. Il est donc nécessaire de réfléchir aux perspectives d'évolution, d'anticiper les potentielles reconversions de ces activités et d'identifier, dès aujourd'hui, les stratégies industrielles à mettre en oeuvre sur les territoires qui seront affectés sur le plan économique et en termes d'emploi par l'arrêt de la production d'hydrocarbures. L'échéance de 2040 n'est pas si lointaine. L'avenir de ces territoires est à repenser et à reconstruire dès aujourd'hui. Pour cela, il nous faut trouver de bons outils. vous avez proposé, dans votre plan Climat, un outil particulièrement innovant pour répondre à ces préoccupations : les contrats de transition écologique et solidaire, les CTE, qui devraient permettre d'accompagner la reconversion des territoires touchés par la sortie progressive des énergies fossiles.

prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l'accompagnement des entreprises et des territoires impactés par la fin progressive des activités d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures, ainsi que sur la reconversion des territoires concernés. Nous souhaiterions

présente notamment le dispositif des contrats de transition écologique et solidaire, destinés, d'une part, aux salariés et, d'autre part, aux territoires concernés. Il expose les différentes modalités possibles de ces contrats, les moyens budgétaires et l'organisation nécessaires à leur déploiement dans le cas d'une stratégie industrielle d'anticipation des mutations liées à la transition énergétique. » Quel est l'avis de ? Cet amendement tend à compléter le rapport prévu au présent article par une présentation des contrats de transition écologique et solidaire. Ces contrats ont en effet été annoncés par le Gouvernement, mais sans précisions, à ce stade, sur les modalités ou les moyens budgétaires qui pourraient leur être dévolus.

Monsieur le sénateur, j'ai effectivement conscience que les

que, « pour tous les salariés dont l'emploi est directement menacé par la transition à moyen terme, comme c'est le cas dans la production d'énergies fossiles, nous mettrons en place des contrats de transition écologique. Ces contrats associeront les parties prenantes- salariés, collectivités territoriales, entreprises, État -dans la recherche d'un objectif commun de reclassement optimal pour les salariés, en utilisant et en faisant évoluer les outils existants.

Monsieur le ministre d'État, lors de l'examen du projet de loi par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, nous avons été nombreux à craindre que l'on substitue à la production nationale d'hydrocarbures des importations d'hydrocarbures non conventionnels, comme le gaz de schiste ou le pétrole issu de sables bitumineux, dont les méthodes d'extraction sont très néfastes pour l'environnement et entraînent le rejet de volumes importants de gaz à effet de serre. Comme je l'indiquais au cours de la discussion générale, il s'agit d'un problème très actuel, puisque, dans le cadre des négociations relatives au CETA,

Cela a conduit les députés à prévoir, à l'article 3 , la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur l'origine des pétroles et gaz importés, ainsi que sur leur impact environnemental. Il s'agit d'une première étape, qui devra permettre d'apprécier la possibilité de différencier les hydrocarbures en fonction de leur bilan carbone sur l'ensemble de leur cycle de vie. Il pourrait être envisagé, à partir des conclusions de ce rapport, de moduler la taxation sur les produits pétroliers en fonction de leurs émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de leur cycle de vie. Monsieur le ministre d'État, quelles actions comptez-vous promouvoir aux niveaux national et européen sur ce sujet ?

La mise en place de la traçabilité proposée par les auteurs de l'amendement, de même que la définition des critères retenus, se heurte aujourd'hui à des difficultés techniques, voire géopolitiques,

Le scrutin est ouvert.

les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

économiques du Sénat a fait le choix de supprimer un article qui permettait d'aller au-delà des symboles en appréhendant la question des hydrocarbures sous un angle plus large que celui de la seule production nationale. de portée limitée, certes, permettait de prendre en compte les activités d'exportation. Ainsi, le Gouvernement se voyait enjoindre de remettre un rapport au Parlement sur les concours de toute nature de l'État en soutien aux activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures hors du territoire national.

Actuellement, les subventions de l'État destinées aux activités nationales d'exploration, d'exploitation et d'acheminement d'hydrocarbures, notamment de pétrole et de gaz, sont distribuées sous forme d'exonérations de taxes ou par le financement direct d'infrastructures, comme les terminaux méthaniers et pétroliers. La France a dépensé 395 millions d'euros par an entre 2014 et 2016 en financements internationaux pour la production de combustibles fossiles et l'exploitation d'infrastructures électriques. Depuis plus de trois ans, 22 % de ces projets concernent des activités d'exploration et d'extraction d'hydrocarbures. Or, comme l'exposé des motifs l'indique, le présent incitera les investisseurs à orienter leurs investissements à court et moyen terme vers d'autres pays. Il n'est donc plus souhaitable que l'État continue de financer ces dépenses.

Il vise à rétablir la demande de rapport sur les subventions accordées par l'État aux activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures à l'étranger. Ce rapport permettra d'étudier la cohérence de la politique de la France en matière d'énergies fossiles et de prendre les mesures qui conviennent.

qui a été adopté par les députés et supprimé par la commission des affaires économiques du Sénat. Nous proposons que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les concours de toute nature de l'État en soutien aux activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures menées hors du territoire national. Nous savons que les soutiens aux énergies fossiles sont extrêmement importants et se chiffrent en centaines de milliards d'euros. Ce projet de loi vise à mettre fin progressivement à l'exploration et à l'exploitation des mines d'hydrocarbures à l'horizon de 2040. Il s'agit bien évidemment de donner l'exemple ; ce texte est pionnier en la matière, dont nous nous félicitons. Reste que l'effort doit également porter sur le recensement des aides et des subventions destinées à l'industrie pétrolière hors de nos frontières. est le sens de cet amendement, dont l'adoption permettra de porter haut l'ambition du Gouvernement, qui remettra au Parlement un rapport recensant toutes les aides destinées au secteur pétrolier. C'est une question de transparence.

n° 88. En cohérence avec l'esprit du projet de loi, qui vise à restreindre le développement des hydrocarbures fossiles dans les limites des possibilités dont dispose le Gouvernement français,

? L'amendement n° 28 rectifié tend à supprimer tout concours direct de l'État à l'exportation des activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures. des dispositions du présent projet de loi se traduira déjà, à terme, par la suppression de 1 500 emplois directs et de 4 000 emplois indirects dans le secteur de l'exploration-production sur le territoire national.

national que la commission a supprimé au motif de la faible portée opérationnelle d'une telle disposition. Par cohérence avec la position de la commission, j'émets un avis défavorable.

Gontard, sur l'article. L'article 3 prévoit la mise en ligne en de l'ensemble des demandes de titre minier en cours d'instruction et des titres en cours de validité. Il s'agit d'un élément de transparence bienvenu. à l'Assemblée nationale ont permis d'aller plus loin, en indiquant que ces informations devront être assorties d'une carte présentant le périmètre de ces titres sur le territoire national. C'est une bonne chose. renforcement de la transparence est d'autant plus justifié que ces informations étaient accessibles jusqu'au 31 décembre 2015, avant que le ministère ne les retire de son site internet dans le cadre d'une refonte de celui-ci. Aujourd'hui, il ne reste en ligne qu'une simple liste des permis en cours de validité au 1 juillet 2017. Nous considérons qu'il est nécessaire d'aller plus loin. Il convient non seulement de rendre publique la carte des périmètres des titres miniers, mais également d'éditer un bulletin mensuel d'information. Ce bulletin rendra publics les titres miniers déjà attribués et les dossiers en cours d'instruction, avec le lien vers les préfectures. L'intégralité des documents requis pour l'enquête publique et des décisions administratives d'autorisation de travaux sera accessible. Il convient également de rendre publiques les références aux décisions de justice concernant les concessions et les arrêtés de rejet ou de refus relatifs aux permis et concessions. Par ailleurs, toujours dans un souci de transparence, nous estimons nécessaire que le Gouvernement communique la liste récente des recours et des jugements en dernière instance déjà prononcés. Il me semble qu'une communication de ce type permettrait, monsieur le ministre, d'instaurer un climat de confiance, notamment avec les associations environnementales. Nous constatons, encore une fois, l'urgence d'une révision du code minier, notamment de sa partie relative à la participation du public. La mise en place d'une véritable transition énergétique, l'adhésion à des pratiques nouvelles ne pourront se faire que dans la concertation, la participation et la transparence. J'ajouterai un mot sur la limite instaurée par la commission des affaires économiques, précisant que « les informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété intellectuelle » du titulaire du titre ne peuvent être rendues publiques. Nous ne voyons pas bien quel usage pourrait être fait de cette disposition et souhaiterions disposer d'informations plus précises sur cette limite,

rapporteur de la commission du développement durable de l'Assemblée nationale, va dans le sens de la plus grande transparence de l'information du public souhaitée par le Gouvernement. 53 rectifié vise à le compléter. La mise en ligne des informations relatives aux demandes de titre minier doit valoir pour toute la durée de vie d'un titre- octroi, prolongation, mutation, extension pour que les informations transmises soient exhaustives. Afin de permettre l'information la plus complète et la plus utile possible, cet amendement vise à mettre également à disposition du public les décisions administratives relatives aux projets miniers en cours. De même, les études d'impact environnemental sont des éléments importants qui permettent une bonne appréciation des enjeux économiques et environnementaux d'un projet minier et relèvent donc de la publication des informations administratives prévues par cet article. La centralisation des informations contribuera à la transparence et à l'accessibilité de l'information sur les projets miniers. Pour atteindre l'objectif de transparence et d'accessibilité des données, il importe également que ces données brutes soient exploitables dans un standard ouvert et librement réutilisable. En outre, leur actualisation devra être relativement fréquente.

informations associées à l'activité minière. Je peux déjà vous annoncer que la carte et la liste des titres miniers en cours de validité et en cours d'instruction ont été publiées, mises à jour, sur le site internet du ministère la semaine dernière.

de travaux miniers- forages, etc. -, qui sont déjà mises à disposition du public par les préfectures sur leur site internet lors de l'enquête publique.

du rapporteur de la commission du développement durable. Il prévoit, dans un souci de transparence, que soient mis en ligne en, dans le mois suivant la promulgation de la loi, l'ensemble des demandes en cours d'instruction de titres d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux, l'ensemble des titres d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux en cours de validité, les caractéristiques principales de ces demandes et titres et une carte présentant leur périmètre sur le territoire national. L'article prévoit également que ces données soient actualisées tous les semestres. Nous avons été alertés par des associations qui, si elles se félicitent de l'avancée en matière de transparence que représente cet article, s'interrogent sur la périodicité d'actualisation des informations devant être mises à la disposition du public. Ces associations considèrent qu'il serait nécessaire que ces données soient actualisées chaque mois, et non tous les semestres. Selon elles, jusqu'à la fin de 2015, l'ancien bureau « exploration-production des hydrocarbures », devenu « bureau des ressources énergétiques du sous-sol », publiait un bulletin mensuel d'information mis en ligne chaque début de mois sur le site ministériel.

les demandes de titre, ainsi que leurs caractéristiques principales. Nous craignons que la disposition adoptée par la commission des affaires économiques du Sénat,

couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété intellectuelle du titulaire du titre ne peuvent être rendues publiques. Ces données relèvent déjà du champ des informations protégées. Par ailleurs, on voit mal en quoi ces éléments, sensibles sur le plan commercial et industriel, seraient de nature à améliorer l'information du public. L'avis de

fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement (n° 21,